relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, afin de mener sa mission d'information sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements.

les événements de ces derniers jours, ce qui est désormais appelé « l'affaire Benalla », et l'onde politique et médiatique qui en a résulté ont provoqué une désorganisation des travaux parlementaires. Je ne vois pas comment les textes en lecture à l'Assemblée nationale pourront être examinés, dans ces conditions, avant la fin de la session extraordinaire. Dans une démocratie, il est des moments où le Parlement a le devoir d'affirmer son rôle de contre-pouvoir institutionnel.

Une fois encore, le rôle du Parlement, particulièrement du Sénat, paraît indispensable, celui d'un contre-pouvoir exigeant, dans le respect de nos institutions mais aussi pleinement dans l'actualité. Je réunirai cet après-midi les présidents de groupe pour organiser la semaine, d'ici à la conférence des présidents, programmée mercredi. D'ores et déjà, le calendrier et le contenu même de la révision constitutionnelle me paraissent devoir être repensés.

Les événements médiatico-politiques de ces derniers jours mettent en évidence des dysfonctionnements majeurs dans l'exercice du pouvoir ; le Sénat ne saurait l'accepter. Rien ne nous est épargné : confusion des pouvoirs, mensonges- pour le moins, manque de transparence -, sentiment d'impunité, commentaires assez surréalistes de certains membres du Gouvernement à la presse ... Ainsi, nous apprenions ce matin que M. Benalla était bagagiste C'est indigne de la République et irrespectueux pour les parlementaires, et pour l'ensemble des Français. Dans cette confusion, plus que jamais le Sénat jouera le rôle qui est le sien, celui de contre-pouvoir, de garant de la continuité de l'État et de législateur.

dans ce désordre, je m'interroge sur la suite de l'ordre du jour de cette session extraordinaire. La conférence des présidents devrait nous éclairer à ce sujet. Je me permets de vous indiquer, monsieur le ministre, que, au regard de l'avancée de l'examen de ce texte majeur qu'est le projet

était détenteur d'un badge qui lui permettait de pénétrer jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On peut s'interroger sur les raisons qui motivaient la possession de ce badge. Devant la pression, notamment celle de l'opposition à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a entendu a entendu l'impossibilité de poursuivre le débat sur le projet de loi constitutionnelle, parce que cette affaire fait, justement, vaciller nos institutions. Que les commissions des lois des deux assemblées se soient dotées des prérogatives des commissions d'enquête et se mettent au travail est une bonne chose. Pour autant, monsieur le président, nous avons besoin d'un certain nombre de précisions. Nous en aurons sans doute cet après-midi, mais je tiens à citer dès cet instant

que l'article 50-1 de la Constitution, qui précise un certain nombre de prérogatives, ne soit pas activé dès maintenant.

il est heureux que les plus hautes autorités de l'État et le Gouvernement se soient enfin rendu compte, durant le week-end, que ce que l'on appelle désormais « l'affaire Benalla » ne pouvait pas être traité d'un revers de main. En effet, nous avons cru comprendre, ce matin, que certains avaient enfin mesuré la gravité de la situation. Il est également heureux que l'on ait compris que les travaux du Parlement ne pouvaient pas se poursuivre comme si de rien n'était et que, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat,

Monsieur le président, à l'heure où le Gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, tente d'affaiblir le Parlement, la presse et les corps intermédiaires, les Français se rendent compte, avec cette affaire, de l'importance de notre assemblée, de l'importance du bicamérisme et du pouvoir de contrôle du Parlement, qui est nécessaire dans notre démocratie. La parole est à M. Didier Guillaume,

d'un homme qui a perdu pied après avoir pris des responsabilités inacceptables et inadmissibles. La commission d'enquête fera ce qu'elle a à faire,

je siégeais encore parmi vous, j'aurais bien évidemment demandé la parole,

au coeur de la République, un élément essentiel de la démocratie et de la représentativité de nos territoires et de ses habitants. Je n'ai donc pas de commentaire particulier à faire sur

du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour mener une mission d'information sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas

ou en perte d'autonomie sous-louant un logement, afin de renforcer la mixité intergénérationnelle et de lutter contre l'exclusion des personnes handicapées.

fondée sur des accords gagnant-gagnant, parce qu'elle permet, d'une part, de donner un logement à des jeunes disposant généralement de ressources faibles et, d'autre part, d'accompagner et de prévenir le vieillissement et de maintenir l'autonomie des personnes âgées. C'est la raison pour laquelle il convient, à mon avis, de donner une base juridique au contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, pour que celui-ci encadre clairement les relations entre les deux parties, notamment concernant la contrepartie financière exigible et l'échange des bons procédés entre la personne âgée et le jeune. Il s'agit surtout de garantir le développement de cette pratique, dans le respect tant des personnes âgées que des jeunes.

d'obtenir des délais et de rétablir le bail à la condition expresse de la reprise totale du paiement du loyer et des charges dès le jour de l'audience devant le juge de l'expulsion. Toutefois, l'article 40 ne prend pas en compte le cas des ménages les plus pauvres en situation de surendettement, notamment à la suite d'une dette de loyer. dette de loyer. Ils seront en effet dans l'incapacité de reprendre le paiement intégral du loyer et des charges, soit parce que le versement de l'allocation logement aura été suspendu du fait de la dette locative, soit parce que les ressources du locataire sont insuffisantes pour reprendre le paiement intégral ou partiel du loyer et des charges.

la reprise intégrale du paiement des loyers et des charges rend constitutionnel le principe introduit par la loi du 6 juillet 1989 sur lequel s'appuie l'article 40 du projet de loi. J'émets donc un avis

Il s'agit de mettre fin à la pratique inhumaine des expulsions locatives qui frappe des familles, des enfants, privés de leur domicile. Cette disposition permettrait, d'une part, d'inciter à la recherche de solutions de relogement adaptées lorsqu'un ménage ne peut pas, ou ne peut plus, faire face au coût de son logement et, d'autre part, d'éviter la multiplication des expulsions locatives frappant des ménages, fragilisés par la progression des dépenses de logement et que le moindre accident de parcours peut faire basculer dans l'exclusion. Les propriétaires ne seraient pas lésés par cette mesure puisque, bien évidemment, comme la loi l'indique, le refus de concours de la force publique leur permet d'obtenir une indemnisation équivalente au loyer et aux charges du logement. les prescriptions internationales en termes de droit au logement, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la convention européenne des droits de l'homme, l'État doit garantir le fait que personne ne peut être privé de son logement en raison de conditions de ressources insuffisantes. Notre amendement tend simplement à garantir ces principes. Outre son objectif de respect de la dignité humaine, il nous semble également en adéquation avec le caractère constitutionnel du droit au logement. Certains d'entre vous opposent à cette mesure la décision du Conseil constitutionnel de 1998 sur la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Nous voudrions clarifier le débat l'inconstitutionnalité d'une telle mesure n'est pas avérée. En effet, si le Conseil constitutionnel s'est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, la rédaction même de cet amendement ne soumet en rien l'exécution d'une décision de justice à une diligence administrative : elle interdit toute décision judiciaire en ce sens.

cette mesure est aussi contre-productive pour le locataire que pour son bailleur. En effet, le débiteur n'aura pas le temps nécessaire pour activer les dispositifs qui pourraient l'aider à reprendre les paiements ou à rembourser sa dette de loyer. Quant au commandement de quitter les lieux, le délai de deux mois pendant lequel l'expulsion ne peut intervenir semble déjà incompressible pour organiser les opérations de la « dernière chance »- reprendre le paiement, saisir le juge pour demander des délais si les circonstances le justifient ou encore saisir différentes instances comme la CCAPEX,

pour permettre la saisine coordonnée des dispositifs d'apurement de la dette locative et organiser le relogement des locataires qui ne peuvent se maintenir dans leur logement. La réduction drastique de ces délais

aux intérêts du bailleur, permet au locataire en difficulté de trouver des solutions afin de régulariser sa situation et, en dernier recours, de rechercher un nouveau logement. Ainsi, le droit en vigueur est plus favorable au paiement de dettes locatives. Pour ces raisons, nous proposons également la suppression de cet article.

Actuellement, la procédure d'expulsion d'un débiteur prend au moins six mois. Nous considérons que la longueur de ces délais pénalise lourdement le bailleur et ne peut que décourager les propriétaires de s'engager

et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 prévoit un transfert du contrat de location en cas de décès du locataire au bénéfice du conjoint ou du partenaire de PACS, ainsi que, s'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis au moins un an, du concubin notoire, des personnes à charge, des ascendants ou descendants. L'article 40 de la même loi précise les modalités d'application de cet article dans le parc social. parc social. La commission des affaires économiques, par l'adoption d'un amendement, a inséré une disposition prévoyant que les bénéficiaires d'un transfert de bail, en cas de décès du titulaire, ne soient pas exonérés de la condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français requise pour l'attribution d'un logement social. est étonnante, parce que ce transfert de bail n'est jamais automatique : il est assujetti à des conditions de durée, soit au moins un an de vie commune, et il concerne un nombre extrêmement limité de personnes, à savoir le conjoint, le partenaire d'un

En conséquence, nous proposons de supprimer l'article comportant cette disposition particulièrement inhumaine et contraire aux valeurs de notre République, notamment au principe de fraternité, qui compte encore en France, comme l'a montré la récente décision du Conseil constitutionnel relative au délit de solidarité. Quel

une clause résolutoire en cas de « non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée La commission des affaires économiques a inséré, par voie d'amendement, une disposition au sein de l'article 40 permettant de considérer que cette clause est réputée écrite dès la conclusion du bail et s'applique donc à tous les contrats en cours. Cette disposition, à effet rétroactif, n'est pas respectueuse de l'accord des parties, alors qu'une telle clause ne permet pas au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation. Elle rend également obligatoire l'introduction de cette clause dans les contrats qui ont été conclus après 2007, alors que les bailleurs avaient la possibilité de le faire.

sans illusions, en effet. La question de la spatialisation de l'hébergement d'urgence n'est pas abordée dans le projet de loi. Pourtant, elle mérite un débat. Le plan départemental d'action pour le logement et et l'hébergement des personnes défavorisées doit définir, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. La loi prévoit que la capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 1 000 ou 2 000 habitants en fonction de la taille de la commune.

fond ? C'est un amendement d'appel, vous l'avez dit vous-même, visant à prévoir un rapport. J'ai l'habitude de répondre le plus longuement possible, mais j'estime qu'il n'y a pas là d'autres observations à formuler.

en permettant de déroger à la procédure d'appel à projets jusqu'au 31 décembre 2022, afin d'inciter les centres d'hébergement d'urgence régis par le régime de la déclaration à rejoindre le régime de l'autorisation, à l'instar des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Ainsi le présent amendement vise-t-il à supprimer la référence aux appartements de coordination thérapeutique, qui ne correspond pas à l'objet du projet de loi. Quel est l'avis de

ainsi libellé : La parole est à M. Alain Fouché. Cet amendement prévoit la remise d'un rapport sur le dispositif expérimental de facilitation de la transformation des centres d'hébergement d'urgence, les CHU, en centres d'hébergement et de réinsertion sociale,

Cet engagement a été tenu, mais il faut que cette expérimentation ne reste pas lettre morte. Il convient donc que le Gouvernement mène, à son issue, une évaluation en vue de sa généralisation et remette en ce sens un rapport au Parlement. Quel est

les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une communauté Emmaüs pour aider les autres. Elles bénéficient ainsi d'un lieu de vie, d'un accompagnement spécifique et mènent une activité tournée vers la solidarité. Depuis Dans le même temps, l'activité menée par les compagnons ou compagnes doit dégager l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des compagnons. Cette approche est ainsi en rupture avec les logiques d'assistanat et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.

au sein du code de l'action sociale et des familles, une nouvelle catégorie d'entité juridique, les OACAS. Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret

Les organismes concernés pourront ainsi contribuer au plan Logement d'abord en développant en toute sécurité juridique des solutions de logement adapté en réponse à des besoins spécifiques. Une circulaire viendra préciser les conditions de mise en oeuvre de cette mesure. La parole est à M.

du projet de loi renforce les moyens de pilotage et d'organisation du dispositif d'accueil et d'hébergement vers l'insertion et le logement destiné à ces personnes.

n° 621 rectifié. Les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, selon le principe posé par l'abbé Pierre « Viens m'aider à aider ».

Si certaines communes vont au-delà de ce qu'impose la loi, il semble important d'augmenter le minimum légal de l'offre disponible sur l'ensemble des territoires concernés. Ainsi, au sein de la métropole du Grand Paris, treize communes concentrent 60 % de l'offre de places d'hébergement existante. Un meilleur équilibre géographique de la répartition des places permettra d'accompagner la logique du Logement d'abord, en intégrant les outils de passage de l'hébergement au logement dans une logique territoriale plus affirmée. Par cet amendement, il est proposé d'augmenter le nombre de places d'hébergement par tranche d'habitants. Quel est l'avis de

de mieux répartir les places d'hébergement. Comme vous, je suis bien conscient que les maires ne se précipitent pas tous pour créer ces places, particulièrement dans la métropole du Grand Paris. La question de l'hébergement à l'hôtel est peut-être la question

les établissements hébergeant des enfants handicapés, les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif, les centres d'hébergement les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les lits halte soins santé et les centres d'hébergement d'urgence. En revanche, certaines structures à vocation sociale et soignante ne bénéficient d'aucun dispositif fiscal. Je pense notamment aux lits d'accueil médicalisés.

qui vise à améliorer la lisibilité du droit s'agissant du régime de TVA applicable aux structures d'hébergement. Mais cet objectif peut être atteint par voie réglementaire, notamment les lits d'accueil médicalisés, ce qui ressort d'ailleurs de l'objet de votre amendement. En outre, s'il fallait en passer par la loi, ce qui ne me paraît pas

l'objectif d'offrir des solutions de logement aux jeunes salariés et aux apprentis en situation précaire, mais le quota de 30 % au bénéfice des publics fragiles répond parfaitement aux objectifs de la politique du logement en zone tendue.

M. Maurice Antiste. Il est proposé que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, ou CRHH, devienne le comité régional de l'habitat, de l'hébergement et de l'aménagement du territoire. Il s'agit d'ancrer les politiques de l'habitat dans les territoires, en lien avec les départements, les agglomérations et les communes. titre des enjeux de gouvernance, le renforcement de la place des régions dans les stratégies régionales de l'habitat est souhaité. Mise à part leur présence dans les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, les régions ne sont aujourd'hui pas reconnues comme des acteurs de l'habitat. Alors que la mise en oeuvre des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mis en place par la loi NOTRe suscite des interrogations sur le rôle futur des régions, un CRHH renouvelé, coprésidé par l'État et la région permettrait de repositionner les régions comme acteur de premier plan des équilibres territoriaux locaux en matière d'habitat.

est à M. Maurice Antiste. L'article 244 X du code général des impôts prévoit un mécanisme de crédit d'impôt destiné à financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer. Ce crédit d'impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations, note étant prise qu'il s'agit d'investissements à long terme, les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de cinquante

Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d'acter, dans la loi, le principe selon lequel ce crédit d'impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux. Quel est l'avis de

dans lesquels cet habitat inclusif peut se constituer. Il s'agit de poursuivre une démarche engagée à l'Assemblée nationale en vue de répondre à une forte demande sociale.

Cet amendement vise à codifier le renvoi à des mesures réglementaires d'application du nouveau titre du code de l'action sociale et des familles relatif à l'habitat inclusif ainsi qu'à procéder à une correction rédactionnelle.

a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services, répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu'alors. Le terme « résidence-services » désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels, maisons ou appartements, équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées offrent des services qui garantissent aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Elles contribuent ainsi, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l'enjeu du vieillissement de la population française ; elles sont de nature à prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées et contribuent à renforcer l'offre de logements adaptés et disponibles. Après avoir mis en oeuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services, qui apportent de vraies réponses au défi du vieillissement et à celui de la qualité de vie des seniors et des personnes à mobilité réduite,

l'habitation dispose que la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département, et ce au moment de l'agrément de l'opération de logement social,

particulièrement intéressante et pertinente. Néanmoins, il est prévu que les locataires devront donner leur accord, ce qui réduit d'emblée, peut-être, la portée du dispositif, puisqu'il faudra chaque année recueillir leur avis et traiter les refus.

annuelle ; en l'état, elle alourdirait les tâches d'enquête des organismes, même s'ils récupèrent les données fiscales sous forme électronique. En outre, vous l'avez souligné, les informations sont particulièrement sensibles. Pour les obtenir directement, le bailleur doit disposer du numéro INSEE des personnes. Or la CNIL accorde à cet identifiant, à juste titre,

possible la transmission directe des informations fiscales. Cela paraît une simplification, mais pose de très nombreux problèmes techniques. En effet, il n'existe pas de système uniforme de gestion des locataires : chaque bailleur dispose du sien

La CNIL, elle, accorde à cet identifiant une protection particulière. Nous avons donc besoin d'approfondir les modalités techniques de mise en oeuvre de ce dispositif pour trouver la voie la plus efficace. Nous sommes totalement d'accord sur l'objectif, monsieur le sénateur Dallier.

pour certaines d'entre elles, leur budget de fonctionnement. C'est évidemment prendre un risque majeur : on garantit ces emprunts pour des décennies ; or, du fait

un contrat d'assurance, sauf pour les étudiants et les apprentis. Cette disposition spécifique était justifiée par l'impossibilité pour ce public d'être couvert par un contrat d'assurance, en l'absence de justification

les dispositions du règlement de copropriété en interpellant directement le locataire occupant en cas de troubles de voisinage ou de mauvais usage des parties communes, par exemple. Dans les faits, il s'avère lourd en termes de gestion. Il est donc proposé d'inverser le dispositif

Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint. Le logement est d'abord le lieu principal où s'exercent les violences et peut également devenir un outil d'emprise pour l'auteur de ces violences : opposition à la vente, mise à la porte, dégradations, accumulation de dettes Ce dernier peut être évincé du logement afin de protéger les victimes de façon temporaire. Beaucoup d'entre elles préfèrent cependant quitter le logement, provisoirement ou définitivement, afin de se mettre en sécurité, souvent avec leurs enfants. Certaines sont alors hébergées chez des tiers, à l'hôtel, dans des CHRS ou dans des services spécialisés. D'autres sont sans abri ou vivent en squat. Toutes doivent chercher un nouveau logement. Qu'elles obtiennent un logement social, une mutation de logement ou un autre type de contrat locatif, ce nouveau « chez elles » pourra être un environnement rassurant et sécurisant où elles et leurs enfants pourront se reconstruire. Pour améliorer les droits des victimes de violences, nous proposions au travers de notre amendement d'étendre le domaine d'application de l'ordonnance de protection à toutes les personnes d'une famille vivant dans le même domicile et de préciser que les violences visées à l'article 515-9 du code civil sont « de toute nature, y compris sexuelles ». En conséquence de cette extension, nous proposions de modifier l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation afin de donner à toutes les personnes protégées par une ordonnance de protection une priorité dans l'attribution des logements sociaux. Malheureusement, comme je l'ai souligné en Nous considérons pourtant que la protection des victimes de violences et d'infractions sexuelles doit continuer à être une priorité pour l'exécutif et le législateur. L'ordonnance de protection est un dispositif qui permet une grande réactivité et une certaine efficacité. Il nous paraît donc important d'offrir à tous les membres de la famille qui résident au même domicile et qui subissent une situation de violence une meilleure protection. Je suis saisi

puisse se voir réclamer par le bailleur le paiement du loyer impayé par son conjoint resté sur place. La disposition du projet de loi prévoyant de mettre fin à cette solidarité va donc dans le bon sens. Toutefois, sa mise en oeuvre risque d'être problématique et, au final, de n'avoir que peu de conséquences concrètes. En effet, il est prévu que la solidarité cesse sous réserve de communiquer au bailleur la copie d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d'une condamnation pénale de l'auteur des violences. Or la production de tels documents induit une procédure longue pouvant durer de nombreux mois, voire plus d'une année, dans le cadre d'une action pénale. La victime de violences se verra donc opposer la clause de solidarité pendant toute cette période.

au moment du dépôt de plainte. Or un dépôt de plainte ne peut pas entraîner de telles conséquences juridiques. Comme cela vient d'être exposé, une plainte peut être

pour l'intégrité des personnes et de la famille ? La Fédération nationale solidarité femmes rappelle que le logement est le principal lieu où s'exercent les violences au sein du couple et qu'il peut devenir un outil d'emprise pour l'auteur de ces violences. Celui-ci peut refuser de quitter le logement ou ne pas payer le loyer. La victime solidaire du paiement des loyers se trouve alors coincée. C'est dans cet esprit que nous avons été conduits à supprimer ce délai de six mois.

de cette nouvelle écriture de la loi. Ainsi, cet amendement vise à supprimer l'alinéa 6 tel qu'il est actuellement rédigé, car il tend à exclure de ce dispositif les victimes de violences conjugales locataires d'un logement non conventionné du parc social, alors que les locataires titulaires d'un bail dans un logement social conventionné pourraient en bénéficier. à étendre le bénéfice de ce dispositif aux locataires victimes de violences et titulaires du bail soumis aux dispositions de la loi du 1 septembre 1948. Quel est l'avis de la commission

On nous dit que l'ensemble du droit de la consommation déborde le seul code de la consommation. Il faut donc que les rapports locatifs soient concernés par l'action de groupe, comme le prévoyait la loi

cite la cour d'appel de Paris : « Il sera surabondamment relevé que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 n'est pas inclus dans le code de la consommation et obéit

C'est pourquoi l'encadrement des loyers est un facteur déterminant de mobilité et de sécurisation des bailleurs ainsi que des locataires dans le parc privé. C'est un dispositif qui a montré son efficacité Il est simplement incompréhensible de le supprimer lorsque le maître mot de l'action du Gouvernement se veut être l'efficacité. L'encadrement limite les abus, améliore le pouvoir d'achat des ménages à un prix quasiment nul pour l'État et constitue la réponse la plus logique à l'argument du prétendu effet inflationniste des APL. Encadrer les loyers, c'est donc agir pour une bonne utilisation des deniers publics. La loi ALUR n'est ni excessive ni confiscatoire après une hausse de quasiment 60 % en dix-sept ans, elle ne vise que les loyers abusifs au-delà de 20 % d'une médiane avec complément de loyer possible. Nous sommes très loin de l'administration du loyer, la loi ne fait qu'imposer un minimum de raison au marché locatif privé. J'ajoute que l'encadrement se situe à un niveau particulièrement élevé, qui exclut de l'accès au logement beaucoup trop de nos concitoyens. Le Conseil constitutionnel en 2014 et les tribunaux administratifs en 2017, à Paris et à Lille, ont validé le principe de l'encadrement. Seule son insuffisante mise en oeuvre est mise en cause. L'encadrement des loyers a donc été annulé pour une question de forme juridique et non de fond. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'abroger l'encadrement et de le remplacer par une expérimentation pour se conformer aux décisions de justice. La prise immédiate d'un décret permettrait à l'État de le mettre en oeuvre progressivement, c'est-à-dire en tout ou partie pour les agglomérations concernées, en se calant sur le déploiement des observatoires locaux des loyers. C'est le sens des amendements que nous défendrons à

de la loi ALUR de 2014 et l'autre réintroduit un dispositif similaire, mais temporaire et optionnel, ne constituent en fait qu'une acrobatie politique visant à inhumer progressivement l'encadrement des loyers. Le projet de loi fait prévaloir un très abscons « droit de propriété » que nous impose la doctrine du libéralisme sur le droit au logement de tous et de chacun consacré par le préambule de la Constitution de 1946. Pour notre part, nous avions soutenu ce principe d'encadrement des loyers avec des réticences. En effet, s'il permet de réguler de manière efficace l'évolution des loyers, il ne permet cependant pas d'en réguler le niveau, ce qui était le propre du dispositif ALUR que cet article vise à supprimer. Pourtant, la cherté du logement en France conduit à des réalités socio-économiques inacceptables : 54 % des ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement parmi eux, 15 % y consacrent même plus de 60 % ! La situation est en constante aggravation, avec une hausse des loyers de plus de 50 % en dix ans sur le territoire français, voire Ce dont nous avons besoin, c'est d'une régulation offensive et pérenne du niveau des loyers, qui serait basée non pas sur le loyer médian comme le prévoyait la loi ALUR-puisque celui-ci incorpore des réalités très différentes du marché locatif -, mais sur un loyer qui reflète les réalités sociales et le niveau de vie des locataires. Pour ce faire, nous devons créer un cadre juridique qui permette aux loyers actuels d'être baissés efficacement et donner une place plus importante aux associations de locataires dans le cadre des recours juridiques. Je le rappelle, à Paris, seulement une centaine de recours ont été déposés pour loyers abusifs durant toute la période de l'encadrement des loyers alors qu'environ un tiers des appartements proposés à la location ne respectait pas le dispositif. En cause, le rapport de force défavorable aux locataires, qui craignent que leur bail soit non renouvelé, leur caution conservée ou les travaux retardés. que, depuis l'abandon de ce dispositif, les prix ont largement augmenté comme en témoigne une étude de plusieurs associations. Encadrer les loyers, c'est protéger les classes moyennes qui ne peuvent pas accéder au parc locatif social, c'est augmenter leur pouvoir d'achat et c'est donc,, relancer la consommation et l'emploi.

Éliane Assassi, sur l'article. L'habitat n'est pas un simple produit de consommation, c'est un droit à garantir : celui d'avoir un toit et de pouvoir se loger décemment. La loi ALUR, certes imparfaite et incomplète, avait au moins le mérite d'apporter une part de régulation pour lutter contre la rente immobilière. En effet, l'investissement dans la pierre est parmi les plus sûrs et les plus rentables ; c'est un objet de spéculation. Pour lutter contre cela, l'État dispose de quelques leviers. Pendant longtemps, le choix fait a été celui de la solvabilisation. Ce choix est aujourd'hui remis en cause par la baisse des APL. Le deuxième levier est celui des aides à la pierre pour favoriser la construction. Avec un budget de l'État plafonnant à 60 millions d'euros, autant dire que ce n'est pas une priorité. Enfin, il y a la réglementation du marché dit « libre » que ce soit concernant les règles de mise en location ou plus activement par un encadrement des loyers. À l'évidence, sur ce point, il existe un consensus entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement toute règle est considérée comme une entrave à la liberté contractuelle. Comme si le locataire ou le demandeur de logement étaient en position favorable face au loueur ! La demande est à ce point déconnectée de l'offre que le rapport entre le bailleur et le locataire est absolument déséquilibré. C'est le pot de fer contre le pot de terre ! Pour cette raison, la loi ALUR avait tenté une amorce de régulation avec un encadrement des loyers, qui a aussi vite été désavoué par le gouvernement Valls, circonscrit à Paris et aux collectivités volontaires. et aux collectivités volontaires. Bien que favorables au principe d'encadrement, nous avions considéré que celui-ci risquait, en l'état, de bloquer les loyers à un niveau anormalement élevé. D'où nos propositions d'un moratoire dans le secteur public et d'un mécanisme dans le privé qui définisse des prix moyens à un niveau plus bas. Quoi qu'il en soit, en supprimant ce dispositif, le présent gouvernement envoie un très mauvais signal.

faire. Des recours ont ensuite été déposés, et les tribunaux administratifs ont annulé le dispositif de Lille, puis celui de Paris, avec les mêmes motifs juridiques. J'ai consulté

de faire confiance aux collectivités et de supprimer la coordination obligatoire entre l'Observatoire des loyers et la mise

parce que des familles subissent des situations intolérables. C'est parfois plus de la moitié d'un salaire qui part dans le loyer